Il s’agit non pas de sanctionner, mais de reconnaître la responsabilité des plus grandes entreprises. Celles ci bénéficient d’infrastructures et d’un cadre public qui soutiennent leur prospérité. En retour, elles doivent contribuer équitablement à financer les besoins essentiels que sont l’éducation, la santé et la transition écologique. Cet amendement est un appel à bâtir une fiscalité moderne et solidaire. Le défendre, c’est contribuer à rétablir l’équilibre entre le pouvoir économique et le devoir social, pour une société plus juste, dans laquelle chacun, y compris les plus puissants, assume sa part de responsabilité.

notre pavillon aérien, déjà confronté à un différentiel de charges sociales estimé à 30 % par rapport aux compagnies non européennes. Dans un contexte de reprise post covid encore fragile, il serait contre productif d’alourdir davantage la fiscalité de ce secteur stratégique. Les amendements

Il s’agit, là encore, d’une proposition de notre collègue Pierre Antoine Levi. L’article 11 instaure une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Si le principe d’une telle contribution peut se comprendre dans le contexte actuel, ses modalités d’application créent des effets de seuil particulièrement brutaux, qu’il nous faut impérativement corriger. En effet, les taux d’application se situent très largement au dessus de la moyenne européenne de 21 %. Le mécanisme de lissage prévu dans l’article sur seulement 100 millions d’euros au delà de chaque seuil est manifestement insuffisant. insuffisant. Une telle brutalité fiscale risque de pénaliser gravement la compétitivité de nos entreprises, notamment celles qui sont en concurrence directe avec leurs homologues européennes. Notre amendement vise donc à donc à élargir ces plages de lissage. Cette modification permettrait une progressivité plus douce de l’imposition, tout en préservant l’objectif de contribution des grandes entreprises au redressement de nos comptes publics. L’amendement

En l’état, une entreprise réalisant moins de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires sera exonérée de la contribution exceptionnelle si elle est indépendante, mais elle y sera assujettie si elle appartient à un groupe fiscalement intégré dépassant ce seuil. Cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de capacité contributive réelle. Elle pénalise simplement le choix de s’organiser en un groupe intégré, qui répond pourtant à des logiques économiques et opérationnelles légitimes. Cet amendement vise donc à rétablir une équité fiscale en exonérant les groupes intégrés

les entreprises qui créent de la valeur en France en choisissant d’y implanter leurs sites de production, d’y recruter et d’y installer leurs collaborateurs sont pénalisées par les modalités de calcul de la contribution exceptionnelle, à l’inverse des entreprises qui réalisent ou transfèrent leurs bénéfices à l’étranger. Concrètement, le coût d’un bien Concrètement, le coût d’un bien produit et créé en France serait alourdi de 10 % par rapport à un même bien fabriqué et conçu dans un autre pays de l’Union européenne. Dès lors, cette surtaxe est contre productive, car elle incite les entreprises françaises à s’interroger, comme cela a pu être le cas par le passé, sur l’implantation géographique de leur production. Pour éviter de tels effets de bord, cet amendement vise à répartir plus justement et plus efficacement

pas cohérent au regard du principe d’imposition des bénéfices, qui permet de tenir compte de la capacité contributive des entreprises. Pour le dire encore plus clairement, ce serait défavorable aux entreprises industrielles, qui ont besoin d’une forte intensité capitalistique

: « Il est institué une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires provenant des opérations ci après définies, réalisés depuis le 1 août 1914, jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suivra la cessation des hostilités. acquittée « par les sociétés et les personnes passibles de la contribution des patentes, dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice normal ». On est complètement dans le sujet

s’applique indistinctement à l’ensemble des secteurs de l’économie. De plus, le critère retenu pour identifier les entreprises redevables est le fait de réaliser un bénéfice

un petit rappel : entre 2011 et 2021, les cent plus grandes entreprises françaises cotées à la Bourse ont versé en moyenne 71 % de leurs bénéfices sous forme de dividendes et de rachats d’actions.

Le budget consacré, 6,7 milliards d’euros sur chacune des deux dernières années, reste loin derrière les montants engagés par ses concurrents directs comparables comme Novartis ou AstraZeneca. Le groupe pharmaceutique français s’est caractérisé pendant trop longtemps par un singulier manque d’ambition dans l’innovation, sinon par une docilité trop prononcée aux exigences de ses actionnaires. » Mais tout va bien

Dans tous les secteurs, que ce soit l’artisanat, la pêche, ou le transport routier, elles leur apportent des services auxquels, seuls, ils n’auraient pas accès. Elles contribuent ainsi aux performances économiques et au maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires. Le sociétariat et la contribution au capital relèvent exclusivement des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative – un associé égale une voix – et la lucrativité limitée – les intérêts aux parts sont optionnels et plafonnés – font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs.

Cette situation n’encourage pas les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. La question de l’autofinancement le renforcement du capital social, plutôt que par l’endettement, est d’une actualité toujours brûlante au regard des taux directeurs des prêts bancaires. Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement et de se développer durablement dans les territoires à proximité de leurs concitoyens. La coopérative leur apporte un panel de services et de solutions mutualisés à la hauteur des exigences réglementaires, environnementales et économiques de notre société. Le rôle économique et social de ce modèle plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires – fournisseurs, clients, Banque

À l’origine, ces labels étaient pensés pour rééquilibrer le jeu du commerce international, qui met sous pression les petits producteurs des pays en voie de développement, afin de leur assurer une juste rémunération. Il n’y a aucune raison que cette logique vertueuse ne puisse s’appliquer aux producteurs français et aux entreprises engagées dans une démarche responsable.

Pour éviter l’augmentation du coût du crédit des sociétés qui sont déjà en difficulté financière, nous proposons, par le présent amendement, de ne pas limiter la déduction des intérêts dus aux créanciers qui participent à une restructuration financière et qui deviennent actionnaires dans le cadre d’une procédure collective par le taux maximum fiscalement déductible du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.

aux associés ont pour but que les associés soient rémunérés par les intérêts normalement déductibles du résultat imposable. Cette limitation n’est pas applicable aux intérêts rémunérant les créances de nature commerciale détenues par les sociétés.

d’infrastructures de transport au rétablissement des comptes publics, au travers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) introduite par la loi de finances initiale pour 2024. Compte tenu de la création de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises souhaitée par le Gouvernement, à laquelle seront assujettis certains de ces opérateurs, il me semble juste d’éviter aux aéroports français une forme de d’ailleurs ce qu’a tenté de défendre hier notre collègue Vincent Capo Canellas. Cette contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés, calculé sur l’ensemble des résultats imposables, lesquels sont établis sous déduction de toutes charges,

les deux tiers de ces sommes concernent une dizaine d’entreprises. Celles ci sont certes très douées pour la recherche et le développement, mais également pour trouver le chemin de l’optimisation fiscale. Nous proposons de plafonner cette déduction fiscale à 20 millions d’euros.

vise à encourager les investissements en recherche et développement en France. Cependant, il présente plusieurs limites qu’il est important de corriger. Premièrement, il faut plus d’équité entre les entreprises. Aujourd’hui, ce sont surtout les grandes entreprises

Deuxièmement, il faut maintenir l’attractivité pour la recherche et développement. Même avec un plafond, le taux réduit de 10 % reste très avantageux. L’outil continuera d’attirer les investissements en recherche et développement et à encourager l’innovation en France, tout en étant mieux encadré.

que sur une fraction infime des plus values qu’elles réalisent lorsqu’elles revendent des parts de sociétés dans lesquelles elles ont investi. Cette exonération colossale profite essentiellement aux holdings patrimoniales et aux grandes fortunes qui les détiennent. La France est à l’euro près, n’est ce pas ? Chaque dépense de l’État doit être justifiée, orientée vers l’amélioration du bien collectif : voilà ce que nous disons depuis le début de l’examen en 2019, Éric Woerth, alors président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, estimait déjà que cette niche fiscale coûtait 5 milliards d’euros par an à l’État.

Cette somme pourrait permettre de renforcer nos services publics, d’investir dans la transition écologique, un domaine où de nombreux efforts sont nécessaires, ou encore de soutenir les collectivités territoriales. Nous y reviendrons bientôt. pourrait financer les politiques publiques essentielles pour le bien commun. Certaines voix s’élèveront sans doute pour dire que cette niche encourage l’investissement dans l’économie. Mais soyons clairs : les chiffres et les faits montrent que, pour l’heure, elle n’a absolument pas l’effet escompté, et cela dure depuis vingt ans. Il est difficile d’imaginer qu’il en soit autrement demain. Au contraire, cette niche encourage un capitalisme prédateur, tourné vers le court terme et la maximisation des profits, qui ne se soucie pas des conséquences sociales, économiques et environnementales. Pour mettre fin à cette injustice fiscale, nous proposons donc purement et simplement de supprimer

Cette subdivision matérialise la décision de gestion de l’entreprise de soumettre irréfragablement lesdits titres au régime des plus et moins values à long terme. La décision de gestion de l’entreprise serait ainsi opposable tant par l’administration fiscale, en cas de plus value, que par le contribuable, en cas de moins value.

je vous remercie

L’amendement tend à instaurer un taux majoré d’impôt sur les sociétés, porté à 30 % dans plusieurs cas spécifiques, lorsque certaines grandes entreprises ne respectent pas leurs obligations sociales et sociétales. Ces dispositions visent à sanctionner, mais surtout à inciter à un comportement exemplaire en matière d’égalité et de responsabilité sociale. Tout d’abord, l’amendement vise les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et dans les instances dirigeantes. Ensuite, nous proposons d’appliquer ce taux majoré aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales d’employer des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total. En outre, nous proposons de sanctionner les entreprises dont les pratiques salariales entraînent des écarts de rémunération excessifs. Enfin, ce taux majoré s’appliquerait également aux entreprises qui ne respectent pas les principes élémentaires de responsabilité sociale et sociétale, tels qu’un objet légitime et une gouvernance au service de l’intérêt commun. Mes chers collègues, cet amendement vise non pas à stigmatiser les entreprises, mais à les inciter à s’engager davantage pour l’égalité, la diversité et la justice sociale.

Le salarié ne pouvant être empêché d’utiliser son vélo de fonction en dehors de ses trajets domicile travail, la mise à disposition de vélos par les entreprises constitue bien un avantage en nature. Or l’Urssaf a précisé que cette une exception en n’étant pas soumise à cotisations sociales. En outre, je propose de préciser les montants défiscalisés par l’État : non pas 25 % du prix total de la mise à disposition de vélo, mais 25 % de la part minimale de 70 % imposée aux entreprises pour pouvoir bénéficier de la réduction fiscale, permettant ainsi une économie fiscale à l’État. En effet, tous les employeurs considèrent que le vélo sera utilisé pour un usage personnel à hauteur de 30 %, qui correspond au coût du vélo pris en charge de cet amendement permettrait donc d’aligner le texte fiscal sur le texte social, en actant que 70 % de la prise en charge est bien gratuite pour l’usage professionnel. Il est primordial de clarifier la situation auprès d’entreprises qui pourraient avoir des réserves

Cet amendement a pour objet de prolonger la réduction fiscale existante pour donner plus de visibilité aux entreprises mettant à la disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction. En effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais supportés, jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’elles mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos. Or la réduction d’impôt est allouée pour des contrats de location d’une durée minimale de trois ans. De ce fait, les entreprises désirant mettre à disposition de leurs salariés une flotte de vélos après le 1 janvier 2025 et bénéficier

d’abord, la doctrine fiscale indique expressément que les vélos mis à disposition peuvent être utilisés pour d’autres trajets professionnels ou privés.

En effet, ce dispositif fiscal ne cible pas suffisamment les filières industrielles dites vertes œuvrant pour une économie décarbonée, telles que l’industrie ferroviaire.

Les opérateurs français soulignent que ce prélèvement touche de façon non négligeable leurs investissements – ils ont versé 3 milliards d’euros entre 2009 et 2022 –, sans raison valable, puisque la finalité initiale du

ont étendu leur influence sur tous les pans de l’économie ; de fait, nombre de commerces dépendent aujourd’hui de leur placement en tête d’une page Google, du réseau logistique d’Amazon ou encore de leur réputation sur Facebook. Ces plateformes n’exercent donc plus sur un marché, elles sont devenues un marché en soi

le rendement s’est élevé en 2023 à presque 700 millions d’euros, ne concerne que les grandes entreprises du secteur numérique qui réalisent un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros

il est adopté,

qui aurait un impact direct et considérable, tant sur leurs conditions de travail que sur leur protection sociale et, par voie de conséquence, sur les comptes sociaux. Comme il n’a pas encore réussi à convaincre le Gouvernement de changer de position sur ce sujet,

vous constatez un problème relevant du droit du travail et vous le résolvez… en créant une taxe ! C’est magique

au moment de la reprise économique post crise sanitaire. Les chiffres sont déments. Entre 2017 et 2022, le chiffre d’affaires de cette entreprise a quadruplé, le résultat d’exploitation a été multiplié par

(CMA CGM) – je ne la citerai qu’une fois – ne peut servir de caution au Gouvernement pour protéger toutes les autres entreprises, qui réalisent elles aussi des profits indus.

Gouvernement prétendait défendre les armateurs européens contre la concurrence étrangère et éviter l’exil fiscal par usage de pavillons étrangers. Or depuis plus de vingt ans, cette la part des navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne a décroché par rapport à l’évolution de l’ensemble de la flotte mondiale : +3,4 % entre 2017 et 2022, contre +7 %., ce dispositif a permis aux compagnies de transport maritime

En une seule année, le coût de cette niche, troisième dépense fiscale du pays, a donc augmenté de près de 50

quelques données : le chiffre d’affaires du numéro trois mondial du secteur a bondi de 33 % en un an, à près de 75 milliards de dollars, grâce à pas moins de 21,7 millions de conteneurs transportés. Le prix de ces a flambé sous le double effet de la reprise économique mondiale après la crise sanitaire et des embouteillages de navires dans les grands ports mondiaux, accroissant le phénomène de rareté. Les

ait initialement été conçu pour protéger les armateurs européens de la concurrence étrangère, il est désormais nécessaire de mieux encadrer la fiscalité de ces entreprises, pour qu’elle reflète davantage la réalité de leurs profits.

comme les reports en arrière des déficits, ne seront imputables. Cette mesure a donc pour objectif de garantir une contribution fiscale plus équitable des entreprises de fret maritime, en adéquation avec leur capacité financière réelle.

Il nous paraît équilibré, et cela pour deux raisons. D’une part, il vise à associer plus justement ces entreprises au redressement des finances publiques, alors qu’elles ont engrangé ces dernières années des bénéfices importants, liés à la conjoncture économique. D’autre part,

Nous pensons que l’on doit être imposé là où l’on produit la valeur et que le pays pollué doit percevoir une compensation raisonnable. Lorsque, chaque été, la moitié de la flotte mondiale de grands yachts se réunit sur la Côte d’Azur, ce ne sont évidemment pas les milieux aquatiques britanniques ou panaméens qui souffrent ! Le gouvernement Le gouvernement estimait d’ailleurs, en 2023, que le coût de la dégradation du milieu marin pour la façade méditerranéenne et pour l’ensemble des dispositifs de gestion du milieu marin

efforts de la part de nos concitoyens, que nous leur demandons de réduire leur consommation énergétique, de limiter leurs déplacements et de rénover leurs logements, comment justifier que, dans le même temps, certains puissent continuer à utiliser des yachts aux émissions absolument démesurées ?

Pour vous donner une idée, ce volume est supérieur à l’empreinte carbone annuelle moyenne d’un Français, qui s’élève, elle, à 4,4 tonnes de CO2.

permettant aux navires de transport de marchandises et de passagers d’utiliser des énergies propres. Il s’agit du dispositif de suramortissement vert, qui a été modifié à l’occasion de la loi de finances pour 2024 et qui doit s’éteindre au 31 décembre de

et, donc, d’attenter à la compétitivité de nos armateurs, mais de plafonner son bénéfice à 500 millions d’euros. Au delà, le taux normal d’impôt sur les sociétés s’appliquerait. On en a débattu tout à l’heure, oui, cette niche fiscale a une utilité, particulièrement pour la multitude d’armateurs propriétaires de quelques bateaux

le différentiel est beaucoup trop important. Et pour nombre d’autres entreprises et secteurs d’activité qui ne bénéficient pas d’un avantage aussi exorbitant, c’est totalement incompréhensible. Tout en préservant leur compétitivité,

de manière significative aux émissions mondiales de CO2. Pour corriger cette distorsion et encourager la transition écologique, nous proposons d’introduire un malus écologique pour les navires les plus polluants,

dans le secteur maritime, tout en préservant la compétitivité des entreprises qui s’engagent activement dans la transition énergétique.

qui disposent d’une implantation en France est une bonne nouvelle. Nous avions soutenu le gouvernement précédent sur ce sujet. L’amendement que je vous propose a été adopté par l’Assemblée nationale. Il vise à faire de la France la nation la plus ambitieuse sur cette nouvelle imposition. Il est clair que le dispositif international adopté va favoriser la convergence des taux d’impôt sur les sociétés des différents pays participants.

Le présent amendement propose de remplacer le taux minimum provisoire de 15 % en 2025, prévu par la loi de finances pour 2024, par un taux minimum provisoire de 23 %, puis de 25 % dès 2026. Ce dernier taux s’alignera ainsi sur les taux d’impôt sur les

dû à raison de la sous imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance. Il s’agit, notamment, de simplifier et de sécuriser le recouvrement de cet impôt.

La plupart des grandes places financières ont opté pour que les fonds d’investissement ne soient pas concernés, comme le prévoit bien la règle de l’ODCE. La France n’a pas choisi cette voie, créant un fort désavantage compétitif pour la place financière française.

Aujourd’hui, le régime des captives permet de constituer des provisions lors des années de faible sinistralité pour être en mesure de faire face à un exercice déficitaire à la suite de survenance de sinistres au cours des années antérieures.

présent amendement vise à réduire le coût du transfert de risque par la création d’une nouvelle provision pour les sociétés d’assurance et de réassurance. Je tiens à préciser que ce dispositif existe déjà dans d’autres pays européens. Nos compagnies françaises se tournent d’ailleurs vers l’étranger, puisque, aujourd’hui, 8 sociétés d’assurance

l’élargissement qui est proposé ici représente un coût substantiel pour nos finances publiques, et il faut être attentif au risque que cet outil soit mobilisé soit mobilisé pour des opérations d’optimisation fiscale par certaines de ces entreprises. On peut également s’interroger sur l’allongement de la durée

en 2025, un rapport au Parlement sur les résultats effectifs du nouveau dispositif français, notamment de la provision pour résilience. Je pense que ce rapport

une demande de retrait.

Il tend ainsi à limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères établies dans des pays hors UE. Le dispositif proposé consiste donc à limiter l’actuel régime des sociétés mère fille aux pays de l’Union européenne européenne et à remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédit d’impôt plafonné.

pour lever les freins à certaines transformations en Scic. Pour rappel, les Scic sont des sociétés qui sont formées autour d’un projet coopératif d’intérêt collectif, qui combinent une gouvernance multipartite, souvent un ancrage local, une lucrativité limitée

à 10 %. On voit bien que c’est par les dividendes que les patrimoines sont accumulés et que cela permet

ne différencient pas les dividendes placés indéfiniment dans une holding à des fins d’optimisation des remontées normales de dividendes entre les filiales et la société mère. Leur risque juridique découle des taux prévus, qui sont sont particulièrement élevés et qui risquent d’être contraires au droit européen. Celui ci impose qu’une société mère puisse retrancher de son bénéfice imposable, au titre de l’IS, les remontées de dividendes provenant de ses filiales.

Par cet amendement, notre collègue Pierre Antoine Levi nous propose d’insérer un article additionnel visant à revaloriser le seuil d’application de la contribution sociale de solidarité des sociétés d’euros à 25 millions d’euros. Ce seuil, fixé en 2016, n’a jamais été revalorisé, malgré une inflation cumulée de plus de 10 % sur la seule période 2022 2024. Cette situation conduit à un élargissement mécanique de l’assiette, touchant de plus en plus de PME, qui représentent, aujourd’hui, 60 % des redevables. Dans un contexte économique marqué par la hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et des taux d’emprunt, il est crucial d’ajuster ce barème. Cette revalorisation permettrait de préserver la compétitivité de nos PME et ETI,

à l’absence de plan de sauvegarde dans les cinq années suivantes. Ce crédit d’impôt mobilise des moyens très importants : la dépense fiscale atteindra 70 millions d’euros en 2025. D’après l’étude d’impact du projet de loi de finances pour 2024, ce crédit

en matière industrielle, tutoyant les 150 millions d’euros par bénéficiaire, voire 200 millions d’euros à 350 millions d’euros dans les régions ultrapériphériques. Il s’agit donc ici de créer une contrepartie à ce déploiement d’argent public à l’intention des entreprises.

Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI), il convient de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) du dispositif d’intéressement et de renforcer la pertinence des négociations des branches professionnelles de l’ESS sur ces sujets. L’intéressement représente un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures du secteur, contrairement aux structures à but lucratif assujetties à l’impôt sur les sociétés. Afin de rendre plus incitative la mise en place d’un régime d’intéressement dans l’économie sociale et solidaire, il convient d’instaurer un régime fiscal des accords d’intéressement applicable à la taxe sur les salaires pour les personnes morales à but non lucratif, tout en augmentant le montant de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les structures aux effectifs les plus retreints, la conclusion de ces accords d’intéressement n’étant pas la plus adaptée à leur modèle.

l’État (PGE) pour aider les entreprises à faire face aux différentes crises économiques qui ont été déclenchées par la pandémie et la guerre en Ukraine. Alors que l’échéance prévue par les textes en vigueur

La difficulté concerne particulièrement les petites et moyennes entreprises du secteur, qui sont plus vulnérables face aux problèmes de trésorerie. En parallèle, le nombre de défaillances d’entreprises du secteur continue d’augmenter

présenter l’amendement n° I 476 rectifié . Cet amendement, travaillé avec One Voice, vise à instaurer une contribution spécifique sur l’utilisation d’animaux dans le cadre d’expérimentations scientifiques, afin de financer le développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale. En 2022, quelque 2,2 millions d’animaux ont été utilisés pour des expérimentations en France. Pourtant, 90 % des traitements testés avec succès sur les animaux se révèlent inefficaces ou dangereux pour les êtres humains. Alors même que certaines méthodes alternatives à l’expérimentation animale existent déjà et sont éprouvées, elles ne sont pas toujours utilisées. Par ailleurs, certaines applications n’ont pas encore de méthode de substitution, faute de recherche en ce sens.

forte visant à réduire l’utilisation d’animaux dans la recherche. En effet, selon un sondage Ipsos commandé par l’ONG One Voice et publié en août 2023, quelque 89 % des Français sont favorables au développement de méthodes substitutives à l’expérimentation animale, eux se déclarent défavorables à cette pratique, exprimant ainsi une forte attente pour une évolution vers des solutions de rechange. La France reste l’un des pays européens ayant le plus recours à l’expérimentation

la dépense fiscale associée, dont je rappelle qu’elle approche les 8 milliards d’euros. Cet aménagement de l’assiette comprend trois mesures. la suppression du dispositif « jeunes docteurs », exorbitant du droit commun et dont l’application actuelle aboutit à ce que le montant de l’aide versée à l’entreprise dépasse, parfois,

paramétrique du niveau de prise en compte des frais de fonctionnement. En second lieu, cet amendement tend à fixer à 15 % le taux d’imposition des revenus issus de certains actifs de propriété industrielle, les.

vise à maintenir le taux réduit d’imposition des produits de cession, concession ou sous concession d’actifs de propriété industrielle à 10 %. La compétition internationale est extrêmement féroce en matière d’innovation, notamment

d’améliorer l’efficacité du CIR tout en préservant son intérêt en matière d’attractivité fiscale et d’incitation à l’innovation. Il est établi que l’efficacité de la dépense fiscale est inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation 1 euro de CIR versé aux petites et moyennes entreprises entraîne un accroissement de 1,40 euro des dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises. Pourtant, le CIR bénéficie principalement à ces dernières : les 100 plus gros bénéficiaires, qui sont de grandes entreprises, perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME, qui représentent pourtant 91 % des bénéficiaires,

et des grands groupes. C’est la raison pour laquelle il est proposé de limiter le CIR à la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et, par conséquent, de supprimer le taux de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

les dépenses liées aux brevets, à la normalisation et à la veille technologique. L’économie estimée par le Conseil des prélèvements obligatoires s’élèverait à 250 millions d’euros.

nous proposons d’introduire, à coût constant, un plafond abaissé à 20 millions d’euros de dépenses de R&D accompagné d’une hausse du taux à 40 % de façon à accroître les créances accordées à ces acteurs. Cet ajustement serait selon nous salutaire pour notre croissance et notre capacité à favoriser la création d’entreprises innovantes.

comme l’ont récemment montré une évaluation de France Stratégie, le rapport du CPO précité, ainsi que le rapport de la mission d’information

en 2021, seulement 190 entreprises ont capté 3 milliards d’euros. Selon le rapport précité de

Cet amendement reprend l’une des propositions de la mission d’information sénatoriale sur le thème « Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l’erreur française ».

D’autre part, il n’incite pas les entreprises à aller vers l’innovation écologique, alors même que celle ci est la condition de notre compétitivité dans le monde qui vient. Ce deuxième enjeu n’est pas nouveau : le Conseil des prélèvements obligatoires appelait de ses vœux

du CIR consistant à supprimer la tranche octroyant un crédit d’impôt de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. Selon le Conseil d’analyse économique, cette mesure permettrait d’économiser près de 400 millions d’euros et de financer ainsi le coût du maintien du crédit d’impôt recherche.

vise à supprimer le taux de 5 % pour les dépenses excédant 100 millions d’euros. En second lieu, il convient d’orienter les dépenses de recherche et développement vers l’écologie en s’intéressant à des investissements durables au titre de la taxonomie européenne. Le taux de crédit d’impôt s’élèverait alors à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et à 40 % pour les petites et

Alors que ce dispositif arrive au terme de son bornage temporel, cet amendement vise, d’une part, à le proroger et, d’autre part, à doubler le plafond de dépenses éligibles pour le porter à 800 000 euros.

Ce crédit d’impôt, réservé aux petites et moyennes entreprises, prend la forme d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 30 % du montant des dépenses engagées jusqu’à 400 000 euros. Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif favorise l’investissement dans les innovations qui n’entrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.

pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant pour les entreprises ne disposant pas d’unité de production résidente sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Le CIR est la deuxième dépense fiscale la plus importante pour un coût de 7 milliards d’euros en 2023.